Acte est donné de votre mise au point. Elle sera publiée au et figurera dans l'analyse politique du scrutin. Nous reprenons la discussion du projet de loi,

Cet amendement d'Hervé Maurey vise à prévoir les mêmes sanctions en cas de non-respect de l'obligation en matière de transparence de l'origine des fonds pour la construction d'un lieu de culte que pour celles qui sont prévues en matière de transparence du financement des associations cultuelles, notamment la publication des comptes annuels. à prévoir que toute personne intéressée du ministère public ou le représentant de l'État dans le département où le projet de construction de l'édifice cultuel est localisé puisse saisir le président du tribunal judiciaire pour enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l'association maître d'ouvrage de produire le plan de financement et, le cas échéant, le bilan financier de l'opération. Par cohérence

Nous le savons, derrière cette mosquée, il y a un pays dont on parle beaucoup, à savoir la Turquie. Strasbourg veut édifier la plus grande mosquée d'Europe dans une capitale européenne- quel symbole ! -et ce juste au moment où Recep Tayyip Erdogan met en danger le monde, et particulièrement

mais l'ennemi n'est pas nommé. Cet ennemi, c'est le séparatisme et la stratégie d'infiltration et de déstabilisation menée par des pays étrangers, notamment par la Turquie, depuis vingt ans, en France comme dans le reste de l'Europe. Le but du président Erdogan est de favoriser le communautarisme et d'entraver l'intégration des Français d'origine turque ou, plus largement, de confession musulmane. Il le dit lui-même : « L'intégration est un crime contre l'humanité. » Il souhaite peser sur la vie publique, bref fragiliser la concorde nationale et les valeurs républicaines. Une telle stratégie passe notamment par des réseaux sociaux politico-religieux de plus en plus puissants, du lobbying et des campagnes d'influence à tous les niveaux. Selon différentes estimations, vous le savez,

Cet amendement vise donc à introduire un principe d'interdiction de financement direct des organisations, établissements et lieux de culte par des États étrangers, afin de limiter le phénomène d'influence d'États étrangers sur des lieux de culte précis. Il est ainsi proposé de préciser que tout financement d'un État étranger ne pourra être attribué qu'à une fédération départementale regroupant des associations cultuelles ou, à défaut d'existence de celle-ci, à une fédération nationale. L'État gardera la possibilité de suspendre ou d'interdire un financement qu'il juge contraire à ses intérêts. Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement

de certains cultes et représenter ainsi une atteinte disproportionnée au libre exercice du culte. D'autre part, le dispositif constitue également une entrave à la libre circulation des capitaux, prévue à l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Une telle entrave est d'autant plus problématique qu'elle n'est pas conditionnée à un risque d'ordre public, telle qu'une menace réelle, actuelle, suffisamment grave et affectant un intérêt fondamental de la société.

connaître les fonds étrangers, mais sans forcément les interdire, le dispositif prévu à l'article 35 du projet de loi semble suffisamment solide. Il garantit la pleine information des pouvoirs publics et leur octroie un pouvoir d'opposition, sans qu'il soit besoin de le compléter par une mesure d'interdiction. Pour l'ensemble de ces raisons, la commission est défavorable

Aussi, l'état de ces fonds étrangers devrait faire l'objet d'un document distinct des comptes annuels des associations cultuelles. À partir de ce document, le commissaire aux comptes effectuerait des attestations de type « ressources provenant de l'étranger » ou bien « avantages fournis par une personne étrangère »,

provenant de l'étranger. Il constitue un apport important du projet de loi, qui a d'ailleurs fait l'objet de l'assentiment de la commission des lois, laquelle ne l'a pas modifié. Cet amendement tend non pas à remettre en cause l'équilibre du mécanisme de contrôle prévu, mais à clarifier la cohérence des opérations juridiques constituant un avantage ou une ressource soumise à déclaration. En effet, il n'apparaît pas pertinent de viser les titres de créance qui ne constituent pas une opération soumise à déclaration.

L'article 36 du projet de loi, qui introduit un plafond de dons pour les dons en liquide, semble pourtant manquer largement cet objectif et risque de créer des contraintes injustifiées pour le financement régulier des cultes. C'est pourquoi cet amendement vise à supprimer cet article.

En effet, l'article 36 prévoit d'interdire tout don versé en espèces au bénéfice d'une association cultuelle et dont le montant dépasse 150 euros. Ce dispositif est absurde : comment appliquer cette limitation quand un don est accueilli anonymement au cours d'une collecte ? Il aurait mieux valu aligner les obligations imposées aux associations cultuelles sur le droit commun associatif. À titre d'illustration, le paiement en espèces de certaines créances d'un particulier à un professionnel est autorisé jusqu'à 1 000 euros, selon les dispositions du code monétaire et financier. Les auteurs de cet amendement comprennent les craintes que ces dons en espèces peuvent susciter, notamment en matière de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. Cependant, ils estiment que cette disposition sera totalement inefficace dans cette lutte et qu'il est encore une fois inutile de créer de nouvelles contraintes à l'endroit des associations cultuelles. Par conséquent, le groupe Écologiste Solidarité et Territoires demande la suppression de cette disposition. Madame la présidente, pourriez-vous aller moins vite ? Nous n'arrivons plus à suivre !

lesquels doivent obligatoirement être déclarés lorsque leur montant excède 3 000 euros pour chaque exercice. Quel est l'avis

Ils sont tout en hauteur et peu esthétiques. Dans nos campagnes, ce sont des éoliennes ; dans nos villes, ce sont des minarets. Attaché à nos paysages, à l'architecture française et à l'aspect de nos villes, j'ai pour moi la cohérence. Je ne veux ni d'éoliennes ni de minarets dans mon pays.

se feront près de chez vous, vous finirez par les refuser. Plus globalement, nous parlons ici de préservation de notre environnement visuel et urbain. Si, demain, des minarets et mosquées géantes poussent partout, nous vivrons toujours en république, mais nous ne vivrons plus en France. La France, malgré ce que veulent les militants laïcards, c'est aussi ses villages et ses clochers, et non pas les minarets et les souks ! Si vous voulez les voir, mes chers collègues, je vous invite à traverser la Méditerranée Que des musulmans aient un lieu de culte financé par des fonds privés, pourquoi pas ? En revanche, nous n'avons pas à subir les délires de conquête de ceux qui veulent imposer leur religion à tous. C'est déjà le cas à Poitiers, où une mosquée géante dotée d'un minaret a été financée par le Qatar. Elle porte le nom de Pavé des martyrs, en référence non pas non pas aux soldats de Charles Martel, mais aux soldats de l'Armée islamique. Imagine-t-on un lieu de culte anglican en France porter le nom de Waterloo ou une église orthodoxe porter celui de Bérézina ? Ces mosquées géantes, que certains appellent des cathédrales, ne sont rien d'autre que des symboles de conquête.

vous accepterez de voir ériger des minarets sur notre terre. Vous en porterez alors la responsabilité devant les maires et les Français, qui sont attachés, eux, à l'identité de leurs villes et de leurs villages.

classe, autrement dit d'une amende de 1 500 euros, pouvant être portée à 3 000 euros en cas de récidive, contre 450 euros au maximum dans le droit en vigueur. Cette accumulation de contraintes et d'aggravations des peines n'est pas compatible avec le respect du libre exercice des cultes, que la République doit reconnaître en application de l'article 1 de la loi de 1905. outre, l'aggravation des infractions n'aura aucun effet concret sur la lutte contre le terrorisme et l'islam radical, elle se révèle stigmatisante pour l'ensemble des cultes. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires demande la suppression de

qui était malheureusement tombée en désuétude. Le quantum des peines, tant en matière de contravention qu'en matière d'emprisonnement, était devenu sans lien avec celui qui régit les infractions de même nature qui existent dans le code pénal. Le paradoxe est donc que les infractions à la liberté de conscience et à la laïcité sont actuellement moins réprimées que celles qui touchent aux discriminations et à la haine. fait. Il est nécessaire et cohérent d'unifier les peines prévues afin que la police des cultes puisse retrouver toute son efficacité. Avis défavorable. Quel est

vivons dans un pays de liberté ! Ah bon ? La langue de la France est le français, en vertu de la Constitution, mais nous n'avons jamais interdit à quiconque se trouvant en France de parler dans une autre langue,

Laissons vivre la liberté des cultes dès lors qu'ils respectent la loi ! S'ils ne respectent pas la loi, l'État doit intervenir, point. Tout cela est très simple

et au nom des arguments que j'ai développés, vous feriez bien de retirer cet amendement.

combien j'ai travaillé sur ces questions et combien je suis aux côtés de ceux qui ont choisi la France. Manifestement

les peines prévues à l'article 35 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, la sanction passant d'une peine d'emprisonnement comprise entre trois mois et deux ans à une peine de sept ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Cette aggravation apparaît totalement superflue et abusive aux membres du groupe Écologiste-Solidarité et Territoires. sur la version déposée à l'Assemblée nationale, dans laquelle était proposé le transfert de cette infraction à l'article 24 de la loi sur la liberté de la presse, le Conseil d'État avait émis un avis sévère sur l'alourdissement des peines prévues et sur le principe d'une responsabilité spécifique des ministres du culte. Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires n'est pas favorable au durcissement de la peine proposé par Mme la rapporteure lors de l'examen du texte en commission et demande le rétablissement de l'article 35 de la loi du 9 décembre 1905 dans sa rédaction initiale.

! ... Ils peuvent même constituer un préalable à des actions violentes de nature terroriste. Notre droit est aujourd'hui silencieux sur ce point. Ainsi le présent amendement a-t-il pour objet de créer un délit d'incitation à la haine de la France,

condamnés dans le code pénal les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, la trahison et l'espionnage, l'intelligence avec une puissance étrangère, la livraison d'informations à une puissance étrangère, le terrorisme, etc. On y trouve aussi une définition du mouvement insurrectionnel : « Constitue un mouvement insurrectionnel toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. Sauf erreur de ma part, rien dans notre droit n'interdit l'incitation à la haine de la France. Permettez-moi de citer Clemenceau qui disait

qui la concernent doivent être condamnées

le législateur a jugé bon d'inscrire à l'article 1 le principe de la liberté de conscience. Un siècle plus tard, l'intolérance religieuse et les accusations de blasphème resurgissent dans le débat public. Dans ce contexte, la France doit affirmer que pouvoir quitter sa religion, que ce soit pour se tourner vers une autre ou pour ne pas croire, est une liberté fondamentale. C'est pourquoi cet amendement vise à créer un délit de déni d'apostasie, punissant le fait d'affirmer publiquement que l'apostasie est un crime.

Par parallélisme avec la charte prévue, nous devons inscrire ce principe dans la loi. La liberté de conscience est attaquée un peu plus chaque jour.

? Je comprends l'objet de cet amendement. Il paraît cependant déjà satisfait par le droit existant, puisque les incitations à commettre un crime ou un délit et les appels à la discrimination en raison de la religion

c'est-à-dire que tout fidèle peut présider toute cérémonie. Par conséquent, vous irez chercher le ministre du culte alors que le concept n'existe pas

interdite, mais elle est pourtant bien réelle. La commission s'est déclarée favorable à cette aggravation qui permet de réaffirmer la prééminence du mariage civil sur le mariage religieux.

un peu occulte de l'infraction qui pose parfois difficulté et non la qualification de ministre du culte, qui pour les juges est la personne reconnue comme telle par sa communauté religieuse. Voilà pourquoi il est important de réaffirmer dans ce texte que le mariage civil doit obligatoirement être célébré avant d'organiser

Trop de femmes et de jeunes filles font encore l'objet de pressions religieuses, elles sont encore trop nombreuses à vivre sous la pression d'une captivité conjugale. La captivité conjugale, monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est purement et simplement la continuité du mariage forcé. Car, oui, une cour peut dissoudre un mariage civil, mais pas un mariage religieux. Cela peut sûrement paraître absurde, mais c'est ce qui se passe en l'état actuel des choses. Certes, une femme qui se trouve en captivité conjugale peut divorcer et résilier son mariage civil. Cependant cette résiliation n'entraîne pas celle du mariage religieux. Aussi, certaines femmes sont empêchées de rentrer en France, leur pays d'origine, puisque leur divorce religieux n'a pas été reconnu et que leur famille ne souhaite pas accueillir une femme ayant enfreint la loi religieuse. Dans cette situation, certaines femmes subissent des violences de la part de leur ex-mari ou de tierces personnes. Nous nous devons de garantir aux femmes les droits qui leur sont dus et nous devons refuser ce diktat religieux. C'est pourquoi je souhaite permettre la condamnation de toute personne habilitée à prononcer le divorce dans son culte, lorsqu'elle refuserait d'y procéder alors qu'un divorce civil aurait déjà été prononcé. Nous nous devons voter une telle mesure en tant que pays des droits de l'homme et des libertés. Sachez que nombre de pays et associations à l'étranger nous encouragent en ce sens et comptent sur le soutien du Sénat. Quel

de continuer dans cette voie dans le cadre de l'exécution d'une décision de justice en République française ? Elle n'a plus besoin de l'intervention d'un ministre du culte pour les suites

dans les locaux servant habituellement à l'exercice du culte. Certes, le présent projet de loi viendra enrichir et actualiser de dispositif. Nous observons toutefois une carence. Il apparaît en effet nécessaire qu'une personne condamnée après avoir contrevenu aux dispositions de l'article 26 soit également condamnée à une peine d'inéligibilité. De telles atteintes au principe de séparation du politique et du religieux ne peuvent être sans effet d'un point de vue électoral, au risque que les personnes condamnées soient malgré tout élues à des fonctions publiques, en dépit des condamnations prononcées par les juges.

de cet amendement qu'il s'agirait d'une peine automatique, ce qui n'est pas conforme au principe constitutionnel d'individualisation des peines.

a aussi toujours exprimé avec courage dans le monde son combat pour les libertés. Tous ces facteurs nourrissent la haine des islamistes contre la France et les menaces de nombreux pays étrangers,

et que nous refusions de la mener sur le territoire national. Pour combattre l'islamisme radical, nous n'employons parfois que des outils faibles, lorsque nous ne faisons outils n'étant pas à la hauteur de la menace que nous connaissons, nous devons les renforcer dans ce texte. L'article 43 du projet de loi prévoyait initialement d'interdire à une personne condamnée pour terrorisme de diriger ou d'administrer une association cultuelle, pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

En effet, nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut protéger nos enfants, mais aussi nos adolescents, des intentions malveillantes de personnes condamnées pour des infractions en lien avec le terrorisme. Quel est l'avis de la commission

pour des faits de terrorisme ou d'apologie du terrorisme pour une durée égale à la peine d'emprisonnement, sans être inférieure à dix ans. En effet, les faits mentionnés sont de nature suffisamment grave, à l'encontre de la sécurité de la population et de la Nation, pour que l'interdiction de diriger une association cultuelle soit aussi longue que la peine d'emprisonnement, surtout en cas de libération anticipée. Quel

Je me félicite que vous ayez entendu raison et que vous rejoigniez mes positions. Cet article va dans le bon sens, mais il ne va pas assez loin. Je vous propose donc de l'améliorer quelque peu. L'article 43 prévoit que l'asile soit refusé aux personnes condamnées pour apologie du terrorisme dans leur pays d'origine. Nous n'avons pas à accueillir sur notre sol ceux qui défendent les terroristes, c'est évident. Mais je ne comprends pas pourquoi vous n'étendez pas ce dispositif à ceux qui ont effectivement participé à une entreprise terroriste. Je le redis, même s'ils sont condamnés à mort dans leur pays, nous n'avons pas à les recevoir chez nous. La France est une terre d'asile, mais pas une terre d'asile de fous ! Nos chers collègues de gauche vont comme d'habitude s'émouvoir, eux qui n'aiment rien tant que la défense de l'indéfendable, jusqu'à vouloir sauver la vie de ceux qui veulent nous assassiner. J'ai ce défaut- celui-là au moins, celui-là aussi - : cent terroristes condamnés à mort ne m'empêcheront pas de dormir ; mais pas un jour ne passe sans que je pense aux centaines de victimes de l'islamisme en France. Je préfère un terroriste bien mort à l'étranger à un terroriste bien vivant sur notre sol. Vous allez me dire que ce sont les valeurs que je piétine, que je bafoue les traditions d'asile.

des Français. L'assassin de Samuel Paty était connu pour ses liens avec les terroristes tchétchènes. Et pourtant, la République l'a laissé vivre parmi nous au nom des valeurs. Votre aveuglement idéologique se paie au prix fort, au prix du sang français : depuis neuf ans, les attaques terroristes se succèdent à un rythme effréné, une tous les deux mois. Je refuse, quant à moi, que les terroristes les plus dangereux soient accueillis chez nous, même s'ils risquent la peine de mort. Ils ont pris leurs responsabilités, qu'ils les assument jusqu'au bout, y compris au bout d'une corde si la loi du pays dans lequel ils ont commis leur abomination le prévoit ! Quel est l'avis de la commission ?

L'entrisme est de rigueur. Le djihad s'attaque à tous les territoires de notre Nation, à toutes les institutions- services publics, associations, entreprises ... -et à tous les domaines, qu'il s'agisse de l'économie, de l'enseignement ou du sport ; nous en avons déjà parlé dans cet hémicycle. Afin de protéger d'abord les plus fragiles, c'est-à-dire les mineurs et les jeunes adultes, il apparaît évident d'éloigner les personnes condamnées pour des actes de terrorisme. Le présent amendement vise donc à écarter les auteurs de tels actes de toute fonction en lien avec la direction ou l'exercice d'activités dans le champ du code de l'action sociale et des familles. Il convient de faire de l'interdiction le principe et

de la commission ? Les infractions relatives à l'apologie, en ce qu'elles touchent à la liberté d'expression, font l'objet d'un contrôle vigilant du Conseil constitutionnel.

pour l'essentiel, les dispositions que nous utilisons aujourd'hui. Mais j'ai déjà eu l'occasion de dire qu'un jour viendra- il est même déjà arrivé -où les ennemis de la République sauront lire le code de l'urbanisme

que les chrétiens sont des mécréants, que les femmes ne sont pas les égales des hommes, que l'on se transforme en porc quand on écoute de la musique, toutes joyeusetés que l'on peut entendre et qui sont profondément contraires aux valeurs de la République. Nous pouvons certes poursuivre ces personnes,

L'article 44, mesdames, messieurs les sénateurs, est très important, parce qu'il vise à donner une arme contre un séparatisme qui est en lien direct, non pas avec un attentat terroriste,

Mme Esther Benbassa. L'article 44 dispose, au sein du code de la sécurité intérieure, que le préfet pourra prononcer la fermeture administrative temporaire des lieux de culte dans lesquels des propos haineux sont tenus. sont tenus. Un tel dispositif existe déjà depuis la loi SILT de 2017, et il est inscrit au livre II du code de la sécurité intérieure, à l'article L. 227-1 dudit code. L'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure prévoit également la dissolution des groupements, lorsque des propos constituant une provocation à la haine, à la violence, ou une provocation à la commission d'actes de terrorisme sont proférés. Dès lors, l'introduction de ces nouvelles dispositions dans le code de la sécurité intérieure semble redondante. Cette nouvelle incrimination contribue en effet à rendre la loi pénale, encore une fois, peu lisible et peu accessible, puisque l'ensemble des dispositions sont déjà prévues dans notre arsenal pénal. En outre, les notions d'idées ou de théories

Madame la rapporteure, ? Le Gouvernement souhaite intégrer la nouvelle mesure de fermeture dans la loi de 1905, alors que nous avons préféré qu'elle le soit dans le code de la sécurité intérieure. C'est ce qui nous différencie, monsieur le ministre.

On ne doit pas simplement tenir compte des « idées ou théories », des concepts qui, d'une part, ne correspondent à aucune réalité juridique identifiée et, d'autre part, sont sujets à des interprétations hautement subjectives pour caractériser leur existence ou non. Le dispositif mérite donc

fermeture des lieux de culte ne puisse intervenir qu'après avis et saisine du juge : c'est contraire à la notion même de mesure de police administrative. L'article prévoit par ailleurs toutes les garanties nécessaires en matière de voies de recours et d'intervention du juge dans son alinéa 6. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

alors c'est politiquement, par le débat, qu'il faut les combattre, et non par une interdiction qui évoluera vers autre chose.

souhaite intervenir sur cet amendement après l'excellente démonstration de Jean-Yves Leconte.

Quel sens y a-t-il à sanctionner des idées ou des théories ? Cela n'est pas possible ! On a le droit d'avoir des idées

avec des mots ! Les idées sont incarnées, et je ne vois pas comment on pourrait sanctionner une substance appelée idée qui serait dépourvue de tout langage ... Si vous trouvez une idée

différence d'appréciation avec la commission, puisque l'amendement du Gouvernement vise à rétablir à l'alinéa 3 les mots « ou tendent à justifier ou encourager cette haine ou cette violence

l'alinéa 3 tel qu'il est rédigé après l'examen par la commission des lois : « Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent